Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, comme vous tous, et particulièrement nos collègues de l’Essonne, j’ai appris avec tristesse et effroi le meurtre de Louise, 11 ans, dont le corps a été retrouvé dans la nuit de vendredi à samedi dernier dans le bois des Templiers, à Longjumeau. Bouleversés par le meurtre de cette très jeune fille, face à cet acte de violence à l’égard d’une enfant qui ne demandait qu’à grandir, nous avons tous une pensée émue pour les parents et les proches de Louise, pour ses camarades du collège André Maurois d’Épinay sur Orge, pour ses professeurs et pour tous ceux qui, anonymement, partagent leur chagrin et témoignent de leur soutien. Au nom du Sénat tout entier, je les assure de notre profonde sympathie et je vous invite à observer un moment de recueillement.

J’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses camarades et à ses proches. Je me permets d’associer à ce message mon collègue Jean Raymond Hugonet, sénateur de l’Essonne. Nous partageons leur douleur. Il y a trois semaines, c’était Élias, 14 ans, qui était poignardé à mort à Paris. Monsieur le garde des sceaux, la jeunesse est insouciante et si vulnérable. Nous avons le devoir de la protéger. Ces tragédies ne sont pas seulement des faits divers, mais un fait de société qui appelle une réponse politique forte. Rappelons que cent mille mineurs ont été victimes de violences physiques en 2023. Aujourd’hui, le danger est au coin de la rue, à 500 mètres de la maison, en rentrant du sport, et même dans la cour de récréation. Je pense à ce lycéen de Bagneux dans le département des Hauts de Seine, qui a été poignardé la semaine dernière et a heureusement survécu. survécu. Aucun parent ne devrait regarder son enfant s’éloigner de sa maison, en craignant pour son intégrité. Aujourd’hui, des parents ont recours à des applications de géolocalisation pour surveiller leur enfant Une violence débridée déferle au sein même de nos écoles, qui devraient être des sanctuaires dédiés à l’instruction. Mais je veux aussi attirer votre attention, monsieur le garde des sceaux, sur une autre jeunesse en proie à la violence, qui a perdu ses repères et ne connaît plus aucune limite. Face à ce fléau, il est urgent que la loi change pour prévenir, pour mieux réprimer et, surtout, pour traiter plus efficacement la violence. S’agissant des mineurs, il faut supprimer l’excuse de minorité,

première étape d’une refondation ambitieuse des politiques publiques en faveur de nos territoires. L’objectif était d’apporter des solutions durables aux défis des territoires ultramarins.

Un dialogue approfondi avec les élus et les acteurs économiques devait en garantir l’ancrage local. Près d’un an et demi plus tard, la mise en œuvre de ces engagements semble pourtant souffrir d’un manque de lisibilité.

la vie chère, à la compétitivité économique ou à la continuité territoriale – autant de sujets qui appellent des avancées concrètes et durables. Au moment Au moment où le Président de la République évoque la possibilité d’un référendum en 2025 sans toutefois indiquer les thématiques qui pourraient en faire l’objet, certains de nos territoires ultramarins s’interrogent sur leur avenir institutionnel. Il y a peut être là un sujet de consultation. Monsieur le ministre, pouvez vous nous préciser le calendrier de mise en œuvre des mesures du Ciom ? Comment comptez vous aborder les aspirations institutionnelles émergentes dans ces territoires ?

sont nombreuses. Elles appellent des réponses fortes et suivies dans la durée et une action politique pugnace et constante. Nous avons des urgences : Mayotte – nous en avons déjà longuement

est beaucoup trop lent, nous devons accélérer. C’est d’ailleurs le sens du choix du Premier ministre d’élever ce ministère au rang de ministère d’État : il s’agit de lui donner du poids pour faire avancer les choses. Vous pouvez compter sur ma détermination ; je ne lâcherai rien

ans après le vote de cette loi, force est de constater que beaucoup reste à faire pour parvenir à une société réellement inclusive. Le regard sur le handicap a certes changé : nous avons tous pu mesurer la ferveur entourant les athlètes lors des jeux Paralympiques de l’été dernier,

Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est bien trop élevé et les formations adaptées trop rares. Un tiers des gares SNCF et la moitié des établissements recevant du public ne sont toujours pas accessibles. Sans accessibilité, pas d’emploi, pas de loisirs culturels ou sportifs, pas de vie sociale. Enfin, s’agissant du droit à compensation, autre pilier de la loi de 2005, tout reste à faire en raison du non recours effectif aux droits, des restes à charge élevés, de la complexité des démarches et de la sous évaluation des besoins. L’État se désengage des fonds de compensation du handicap, qui ont pour fonction d’accorder des aides financières aux personnes handicapées, afin qu’elles puissent faire face aux frais restant à leur charge. Dans l’Essonne, l’État réduit son soutien de 4 % à 5 % chaque année

– trop lointain ! Madame la ministre, quelle politique comptez vous mettre en œuvre pour parvenir à des résultats tangibles ? L’État est il prêt à prendre toutes ses responsabilités pour que, vingt ans après, chaque personne handicapée puisse exercer l’intégralité de ses droits et se sentir pleinement citoyenne dans la France d’aujourd’hui

domaine de l’intelligence artificielle, nous avons aussi nos Léon Marchand, nos Teddy Riner, nos Antoine Dupont : je pense à Mistral, à LightOn, à Owkin,

Madame la ministre, hier, au Sénat, nous faisions le bilan des vingt ans de la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Or les 12 millions de personnes en situation de handicap et leurs proches nous font part de l’écart abyssal entre l’ambition affichée par la loi et sa mise en œuvre, et ce malgré de nombreux progrès. La Défenseure des droits indique que la première cause de sa saisine reste le handicap et l’accès aux droits afférents. Cet accès aux droits passe par un guichet unique créé par la loi de 2005, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Alors qu’elles placent l’usager au cœur de leurs décisions, les MDPH ne parviennent pas à gérer les flux croissants de demandes légitimes. Entre 2015 et 2022, il y a eu une augmentation de 40 % des demandes de prise en charge uniquement pour les enfants. Malgré la bonne volonté des personnels qui y travaillent, et que je salue, les MDPH manquent majoritairement de moyens humains pour traiter les dossiers dans des délais et conditions acceptables. Elles sont sous la tutelle de la présidence du conseil départemental. Or les départements, premiers financeurs, sont exsangues et sans autonomie fiscale. Ils ne peuvent être les boucs émissaires des carences de l’État, qui n’assure pas la solidarité nationale ni l’égalité territoriale. Pour autant, la politique du handicap doit rester une politique de proximité, permettant d’ajuster les prestations individuelles de compensation. Outre la complexité des droits et prestations, le parcours du combattant de l’accès aux soins ajoute des freins à l’examen des dossiers. La reconnaissance médicale et le suivi sont autant d’obstacles à franchir.

mais aussi rappeler que chacun des départements détermine la stratégie qui est la sienne en matière d’accueil et d’accompagnement. C’est d’ailleurs un travail tout à fait intéressant à remarquer. Je veux en outre souligner

que ce soit sur l’accessibilité, le logement, l’éducation, l’engagement citoyen, l’emploi. C’est ce que nous aurions dû fêter hier, lors du colloque sur le vingtième anniversaire de la loi de 2005, qui prévoyait d’adapter les politiques publiques pour les personnes en situation de handicap. Cette loi, après celle de 1975, avait créé un immense espoir dans le monde associatif, chez les aidants, chez les personnes en situation de handicap, qui s’étaient, faut il le rappeler, beaucoup impliquées. Certes, et fort heureusement, des avancées ont eu lieu ces dernières années ; mais elles sont, il faut le reconnaître, bien en deçà des objectifs de la loi de 2005. Pour 2025, vous annoncez la gratuité des fauteuils roulants, une avancée significative pour ceux et celles qui souffrent de revenus modestes, d’autant que les personnes en situation de handicap ont un niveau de vie inférieur au reste de la population. Malheureusement, beaucoup reste à faire. C’est un choix politique, un choix financier. Les signes ne sont pas encourageants lorsque vous amputez les crédits de l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées de 50 millions lorsque l’État se désengage au détriment des départements, année après année, alors que les dépenses sociales obligatoires explosent pour l’aide sociale à l’enfance, l’allocation personnalisée d’autonomie et la prestation de compensation du handicap.

Sur le fond, les autoentrepreneurs sont montés au créneau, et nous les comprenons. Beaucoup n’y survivront pas, sauf à basculer dans le travail dissimulé. C’est bien pourquoi le montant des recettes annoncé pour cette mesure a varié du simple au double. Bercy en attendait 800 millions d’euros au départ ; aujourd’hui, on nous annonce 400 millions d’euros. L’administration aurait elle donc anticipé la fraude à La ministre chargée du commerce a annoncé hier à l’Assemblée nationale avoir demandé une étude d’impact. N’est ce pas désavouer une fois de plus les chiffres donnés précédemment ? Sur la forme, l’amendement, adopté au Sénat un dimanche après midi au milieu d’une batterie de secondes délibérations, n’a jamais été à proprement parler débattu par l’ensemble du Parlement.

Sur le fond, au delà de la concertation annoncée, allez vous proposer une étude approfondie de la fiscalité des autoentrepreneurs nous permettant de légiférer rapidement et dans de bonnes conditions ? La parole

Ces derniers jours, les discours et cette pluie éhontée de milliards d’euros tendent à nous faire croire que l’IA sera la solution à l’ensemble de nos problèmes, le nouvel eldorado des investisseurs, le summum du technosolutionnisme qui viendra sauver notre planète. Mais, dans la vraie vie – l’épisode DeepSeek en est l’illustration –, l’IA est une bulle. Les résultats que l’on nous promet depuis deux ans tardent. Il existe aujourd’hui peu de certitudes, mais beaucoup de contraintes. Ce qui est déjà sûr, c’est que l’IA a d’ores et déjà un coût écologique considérable et insoutenable à ce stade. Au delà du coût social à venir, l’IA représente un coût humain

a un impact sur la santé mentale ; elle bouscule la propriété intellectuelle et met en danger nos droits fondamentaux et nos démocraties. Aujourd’hui, seule l’Union européenne propose une réglementation, unique

confirmez vous le soutien sans faille de la France à l’AI Act ? Allez vous œuvrer pour le renforcement de la régulation européenne de l’IA sans céder à la pression des géants de la tech et des grands groupes financiers qui comptent encore se remplir les poches ? En d’autres termes, la France va t elle soutenir le leadership européen face à la vague d’illibéralisme et de dérégulation outrancière

et numérique. Monsieur le ministre, j’associe à ma question les plus de 450 maires, conseillers régionaux et départementaux de Moselle qui appuient ma démarche. À moins de trois mois d’une échéance fatidique, les salariés et les sous traitants de la centrale Émile Huchet de Saint Avold continuent de se battre pour leur avenir. Depuis des mois, nous rappelons que le Président de la République s’est engagé à convertir les centrales à charbon dans le cadre d’une transition énergétique plus juste. À ce titre, un projet de conversion au biogaz a été proposé par l’exploitant du site. Par ailleurs, un projet de production d’hydrogène vert, reconnu d’intérêt commun par la Commission européenne, va faire l’objet d’un financement à hauteur de 20 millions d’euros. Les solutions viables ne manquent pas, mais elles nécessitent un soutien fort de l’État. Sans cela, en avril prochain, c’est un pan entier de l’économie locale qui va s’effondrer. Dans un contexte où les tensions géopolitiques ne cessent de croître, la souveraineté énergétique de notre pays est un enjeu stratégique majeur. La France peut elle se permettre d’affaiblir son indépendance énergétique en sacrifiant Émile Huchet sur l’autel de l’inaction ? Face à cette urgence économique, les cinq sénateurs de Moselle ont déposé une proposition de loi transpartisane pour sécuriser l’avenir de ce site et de ses salariés. Aujourd’hui, je sollicite le soutien du Gouvernement pour faire adopter ce texte dans les meilleurs délais. Monsieur le ministre, allez vous tenir les engagements pris par l’État pour sécuriser la transition du site et donner enfin une perspective claire aux centaines de familles plongées dans l’incertitude ? La parole

Ma question s’adresse à Mme la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Madame la ministre, depuis le début de la semaine, avec le sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle, des bourrasques d’annonces présidentielles soufflent dans les médias. Le Président de la République souhaite que le navire France rattrape son retard en matière d’IA face aux États Unis et à la Chine. Les récentes annonces en rafale suscitent de nombreuses questions. Je ne vous interrogerai pas sur les enjeux de souveraineté nationale que soulève l’annonce de 109 milliards d’euros d’investissements

mais une révolution qui touche dès à présent l’ensemble de notre société, et notamment nos façons d’enseigner et d’apprendre. Aujourd’hui, nous savons que la quasi totalité des lycéens et des étudiants,

dans l’offre de formation continue du ministère de l’éducation nationale. Enfin, nous allons mettre en place un partenariat d’innovation pour développer une IA souveraine, ouverte et évolutive, afin d’appuyer les pratiques pédagogiques de nos enseignants. Vous le constatez, nous nous saisissons

Il risque cinq ans de prison, 75 000 euros d’amende et une peine complémentaire d’inéligibilité. Son crime ? Il a refusé de procéder au mariage d’un étranger en situation irrégulière sur notre territoire ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français Certes, il aurait dû savoir qu’en tant qu’officier d’état civil il ne dispose d’aucun pouvoir pour s’opposer à un mariage, y compris à un mariage impliquant une personne soumise à une OQTF. Il aurait dû savoir que la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne permet pas de subordonner la liberté de contracter mariage à la régularité du séjour. Mais, monsieur le ministre, n’est ce pas le monde à l’envers ?

bien penser les Français d’une telle situation ? Ne faut il pas d’urgence modifier notre cadre législatif ? Et nos maires, qui ne sont pas tous juristes, tant s’en faut, n’ont ils pas droit à une juste protection ? Que compte faire le Gouvernement à cet égard ?

D’abord, sachez que, même si les maires qui sont actuellement convoqués par la justice avaient saisi le procureur de la République au lieu de décider par eux mêmes, cela n’aurait rien changé.

imaginez une cuve qui convient largement aux besoins de ses utilisateurs et que l’on vient subrepticement siphonner pour d’autres usages et d’autres besoins. Un beau jour, inévitablement, elle se tarit. Alors, ceux là mêmes qui l’ont asséchée viennent réclamer aux utilisateurs de quoi la remplir de nouveau. Cette petite fable, c’est l’histoire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Depuis des années, celle ci contribue à la solidarité nationale. Ce sont près de 100 milliards d’euros qui ont été prélevés dans cette caisse, et ce sans aucune contrepartie. Et aujourd’hui, pour la renflouer, l’État vient pomper dans les caisses des mairies, des collectivités et des hôpitaux dans des proportions insensées. Dans le secteur privé, le taux maximal applicable à l’employeur est de 28 %. Pour l’année 2025, le Gouvernement impose aux employeurs C’est déjà considérable, mais ce n’est que le début, car ce taux doit grimper jusqu’à 43,65 % en 2028. Par exemple, la ville de Cognac, en Charente, a une masse salariale de 6 millions d’euros.

La parole est à Mme Annick Petrus, pour le groupe Les Républicains.

Avec un taux de criminalité cinq fois plus élevé que dans l’Hexagone, Saint Martin est confrontée à une insécurité croissante nourrie par le narcotrafic, la circulation illégale des armes et une délinquance de plus en plus précoce. Entre fusillades, braquages et agressions, la population est inquiète et l’image de notre territoire se détériore.

Saint Martin subit, entre autres, une criminalité importée, alimentée par les trafics de drogues et d’armes qui transitent par la Caraïbe. Sans un engagement accru de l’État en faveur d’un renforcement de la coopération sécuritaire avec l’ensemble des États de la région, ce phénomène risque de s’intensifier et d’ancrer durablement la violence sur notre territoire. Il est à noter que les défaillances judiciaires et une réponse pénale insuffisante assoient un sentiment d’impunité. Je sais que la vidéoprotection, qui relève de la compétence de la collectivité de Saint Martin, pourrait constituer un atout supplémentaire dans cette lutte. Hélas ! ce dispositif a été détruit par l’ouragan Irma et son rétablissement n’est encore qu’au stade de l’attribution du marché. En attendant, nous devons faire face à cette insécurité avec les moyens dont nous disposons. Monsieur le ministre, dans ce contexte, quelles actions concrètes l’État entend il mettre en place pour mieux anticiper et enrayer cette dynamique criminelle, qui fragilise Saint Martin et menace la stabilité de l’ensemble de la région ? vous à un renforcement de la coopération sécuritaire et judiciaire avec nos voisins les plus proches de la Caraïbe ? La parole

nos institutions. Alors, que comptez vous faire pour protéger nos tribunaux et ceux qui, chaque jour, contribuent au bon fonctionnement de notre justice ?

Monsieur le garde des sceaux, j’entends vos propos, mais je constate que le Gouvernement contribue à cette ambiance. Ainsi, le Premier ministre reprend à son compte le mythe de la « submersion migratoire pourtant démenti par les chiffres de l’Insee. Le ministre de l’intérieur remet en cause le droit du sol et s’en prend ouvertement à l’État de droit. Enfin, la frénésie législative sur l’immigration joue sur les peurs, au détriment des droits indivisibles des personnes, de la réalité des mouvements migratoires et du respect de l’État de droit, qui garantit à tous dignité, justice et égalité. Rien à voir ! La France a besoin de se rassembler ; votre gouvernement la divise !

madame la ministre, allez vous, dans le Cantal et dans l’Allier comme partout en France et, d’abord, dans la ruralité de montagne, respecter l’engagement national et démocratique, que nous avons pris

égale zéro ! Pas de suppression de postes dans le budget, cela signifie aussi : pas de suppression de postes en solde net dans nos départements

nous avons décidé de faire de la baisse démographique un levier pour la réussite de nos élèves, pour la réduction des inégalités sociales et territoriales, et pour l’accélération des politiques prioritaires que sont pour nous la poursuite du déploiement de l’école inclusive

continuera à répondre au mieux aux besoins des familles. Mes équipes et moi même nous tenons à votre disposition, messieurs les sénateurs, pour examiner plus précisément les conditions d’élaboration de la carte scolaire dans votre département. La parole

à ce jour, la procédure au terme de laquelle sera désignée l’entreprise qui aura la charge de cette mission à compter du 1 janvier 2026 n’a toujours pas été lancée par les services de l’État. De mon point de vue, sans préjuger du résultat de cette procédure, il ne fait pas de doute que le groupe La Poste présente toutes les compétences humaines et les infrastructures nécessaires pour mener à bien cette mission. Il paraît cependant important que les parlementaires puissent avoir un débat de fond sur le service universel postal, ainsi que sur les autres missions de service public confiées au groupe La Poste, notamment sa mission d’aménagement du territoire. Dans un rapport publié en mai 2023, la Cour des comptes estimait que l’accélération de la baisse du volume du courrier, du nombre d’exemplaires de presse distribués et de la fréquentation des points de contact postaux

La Cour des comptes indiquait notamment que, face à ce défi, l’augmentation du montant des compensations ne saurait constituer une solution et qu’une redéfinition profonde du cadre et du contenu de ces missions était nécessaire. Compte tenu des enjeux économiques, sociaux et territoriaux de ces missions de services publics, il est urgent que ces réformes fassent l’objet d’une réflexion dans la perspective de l’échéance de la fin de l’année. C’est pourquoi je souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet majeur d’aménagement du territoire.

fermait définitivement ses portes. Elle était en service depuis 1873, au sein de la même famille. C’est une catastrophe humaine, d’abord : 109 salariés se retrouvent au chômage dans un territoire déjà désindustrialisé, où il ne suffit pas de traverser la rue pour trouver un emploi C’est aussi une catastrophe industrielle : il ne reste plus qu’une sucrerie en Île de France, à Nangis, ville dont j’ai été élu municipal. À l’échelle nationale, c’est la sixième fermeture de sucrerie en six ans ; il n’en reste que dix neuf dans notre pays. Alors, pourquoi ces fermetures ? On connaît les raisons la fin des quotas en 2017, et l’effondrement des prix du sucre et de la betterave. Vient ensuite la crise de la jaunisse, qui a détruit 70 % de la récolte betteravière en Île de France en 2020 et contre laquelle les agriculteurs français sont sans défense. Il existe pourtant une solution

Acte est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle figurera dans l’analyse politique des scrutins concernés. Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande d’intervertir les deux premiers points de l’ordre du jour de notre séance de demain, afin que notre assemblée examine les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi

voix pour et deux voix contre, sur la nomination de M. Philippe Pascal aux fonctions de président directeur général de la société Aéroports de Paris. L’ordre du jour appelle la désignation des dix neuf membres de la commission d’enquête sur les les coûts et les modalités effectifs de la commande publique et la mesure de leur effet d’entraînement sur l’économie française. En application de l’article 8, alinéa 5, de notre règlement, les listes des candidats présentés par les groupes ont été publiées. Ces candidatures seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement. L’ordre du jour appelle l’examen de deux projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation de conventions internationales. Pour ces deux projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié. Je vais donc les mettre successivement aux voix.

au regard notamment du principe d’égalité devant la justice, comportent des inconvénients importants en termes de sécurité juridique pour les justiciables et, plus généralement, pour la bonne administration de la justice justice ». À l’Assemblée nationale, les rapporteurs eux mêmes, pourtant issus de la majorité gouvernementale de l’époque, ont reconnu que le nombre de recours contre les projets concernés était en réalité très faible, et ont admis que cet article répond surtout à une forte attente des professionnels du monde agricole. Dans son avis du 26 avril 2024, la Défenseure des droits se montre, elle aussi, très critique. Elle déclare en effet que « cette réforme contentieuse, motivée par la volonté de sécuriser le déroulement de ces projets, restreint d’une manière disproportionnée le droit au recours de leurs opposants. opposants. […] De tels projets ou politiques publiques sont susceptibles de porter atteinte au droit de vivre dans un environnement sain, garanti notamment par l’article 1 de la Charte de l’environnement. » Nous partageons l’ensemble des réserves formulées par le Conseil d’État et la Défenseure des droits, et nous considérons que cet article répond très maladroitement à la colère des agriculteurs.

L’élevage, c’est une fierté française ! La France est un immense pays d’élevage ! Dire que l’élevage n’attire plus la jeunesse, c’est un contresens, ce n’est pas vrai. Vous ne pouvez pas faire une généralité à partir de ce qui peut s’observer ici ou là. Je connais maints contre exemples d’élevages qui vont bien et qui attirent la jeunesse. Je vous invite à fréquenter un peu plus souvent les comices agricoles, et vous verrez la passion de l’élevage chez nos jeunes… Oui, c’est la réalité ! Ce n’est sans doute pas la vôtre, mais c’est celle que je connais personnellement

proposons de supprimer les alinéas 25 à 27, qui visent à raccourcir les délais de recours d’une requête en référé. Je me permets de vous rappeler l’avis très sévère du Conseil d’État

et en particulier la restriction des possibilités de former un référé pour contester des décisions concernant certains projets agricoles, limite l’accès à un tribunal des opposants à ces projets sans que cette restriction soit justifiée

la cristallisation des moyens, qui interdit de soulever de nouveaux moyens en fin de procédure, une disposition très importante, car les associations qui font des recours contre des projets se saisissent toujours de nouveaux motifs pour faire traîner la procédure

pressés de construire bassines et mégabassines pour chercher ainsi à solder la centaine de contentieux en cours en un seul petit alinéa de ce projet de loi

défenseure des agriculteurs

de deux des trois réformes prévues au présent article et une application à la date d’entrée en vigueur de la loi pour la dernière. Nous ne sommes pas favorables à un tel choix. Au vu des nombreux doutes, critiques et inquiétudes suscités par cet article, il convient de prévoir le décalage de son application dans le temps, afin que des analyses ultérieures puissent réellement

Pour ce faire, il est proposé de renforcer les obligations de motivation et de transparence des avis de l’autorité environnementale, souvent utilisés par des tiers à l’occasion de recours contre des projets de construction ou d’extension d’élevage.

Cela permettrait de faire basculer des exploitations du régime de l’autorisation à celui, moins contraignant, de l’enregistrement.

a allongé la durée de consultation du public d’un mois à trois mois, et introduit deux réunions publiques aux frais et en présence des porteurs de projet. Or ces nouvelles modalités ne sont pas du tout adaptées à des installations dont les porteurs de projet, en entreprise familiale, ne disposent pas des moyens financiers et humains dédiés et sont très exposés du fait de la proximité entre leur lieu de vie et leur lieu de travail. Les deux réunions publiques ajoutées par la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte représentent un frein supplémentaire pour le développement de nouveaux projets. Cela va à l’encontre des objectifs de renouvellement des générations en agriculture et de simplification

au lieu du régime actuel d’autorisation, pour les élevages soumis à la directive IED. Tant que la révision de la directive IED ne sera pas applicable avec la mise en œuvre des futures règles d’exploitation uniforme pour les élevages de 2026, une telle proposition est incompatible avec le cadre

je le retire,

Ces attestations ont été conçues pour les industries et, plus généralement, pour les activités susceptibles d’endommager les sols durant leur période de fonctionnement du fait de l’utilisation et de la manipulation de produits chimiques et toxiques.

d’élevage. Les dispositions du code de l’environnement qui organisent la cessation d’activité pour les ICPE « élevage » soumises à déclaration prévoient que le site doit être mis en sécurité. Les enjeux étant identiques pour les régimes d’autorisation et d’enregistrement, la procédure de cessation d’activité pour les élevages relevant de ces régimes doit être calquée

aux phénomènes électriques et électromagnétiques en raison de leur proximité de plus en plus importante avec les réseaux de transport et de distribution d’électricité, du développement des parcs éoliens ou photovoltaïques, et du développement d’antennes relais de téléphonie mobile.

des émissions de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, de la chaleur, de la radiation, de la création de nuisances, de l’élimination et de la valorisation des déchets, ou encore des risques pour la santé humaine,

notamment les prescriptions qui leur sont applicables. Les exploitations agricoles sont de très petites entreprises, à caractère familial. Leur activité est fondée sur la gestion du vivant. Tout cela les distingue des activités industrielles. Il est donc nécessaire de prévoir des dispositions adaptées à ces spécificités, et proportionnées à l’impact sur l’environnement de ces exploitations et aux moyens dont disposent les agriculteurs, qui ne sont pas comparables à ceux de l’industrie.

Les exploitants agricoles qui souhaitent réaliser une construction doivent, en vue de l’instruction de leur dossier de permis de construire, faire appel à un architecte pour définir le projet architectural de leur future construction. Ce recours obligatoire à un architecte, outre qu’il a un coût pour les éleveurs, complexifie considérablement la réalisation de leurs projets. Actuellement, peu de projets de bâtiments agricoles sont dispensés du recours à l’architecte,

la déclaration des ICPE, qui est pourtant dématérialisée, n’aura plus lieu. L’encadrement sera alors le fait des dispositions du règlement sanitaire départemental,

tant pour les chiens que pour ceux qui les entourent. Il faut bien avoir conscience que les chiens ne sont pas des dispositifs de protection qu’il suffit de multiplier pour renforcer la sécurité d’un site. Ce sont non pas des caméras que l’on place ici ou là, mais des êtres vivants qu’il convient d’accompagner si l’on veut qu’ils

être exonéré du respect des exigences fixées par les textes législatifs relatifs à la protection de l’environnement, en particulier le principe de non régression de la protection de l’environnement posé par le code de l’environnement. Le Conseil d’État constate que les dispositions en cause sont dépourvues d’utilité et propose en conséquence de ne pas les retenir. Pour le dire différemment, on continue avec ce texte d’écrire le droit d’une manière tout à fait curieuse, contrairement à ce qui fait la réputation de notre assemblée. De plus, si des exceptions au principe de non régression, fussent elles applicables, sont créées pour certains secteurs, il deviendrait injuste de les refuser à d’autres.

Une éleveuse du Vercors m’a raconté que, dans les territoires où les collectivités locales n’assuraient pas suffisamment la médiation de son activité, sa vie personnelle devenait très complexe. Elle m’a dit recevoir des dépôts de plainte pour des peurs, des pincements, des chiens qui se baladent dans les jardins. Elle a perdu 10 % de ses 60 hectares

s’était fondé sur la non protégeabilité du territoire. Le premier arrêté préfectoral contesté a été pris pour un troupeau reconnu par le préfet comme non protégeable.

Guillaume Gontard. Cet amendement vise à créer une obligation d’information sur les formations existantes pour les propriétaires de chiens de protection. Il s’agit, j’y insiste, d’une obligation d’information qui incomberait aux éleveurs et éleveuses canins, et non pas d’une obligation de formation pour les éleveurs ovins qui acquièrent un ou plusieurs chiens.

privées et associatives soit bien porté à la connaissance des éleveurs pastoraux. Ces formations de dressage sont fort utiles et contribuent souvent à diffuser également une information juridique sur les obligations des propriétaires de chien, ce qui leur permettra de se conformer aux conditions nécessaires pour bénéficier de la présomption que nous venons de voter à l’article 16.

ou lynx – est éclatée entre plusieurs groupes de travail, chacun dédié à une espèce. Le problème est que certains acteurs, notamment les représentants du monde agricole et pastoral, ne sont pas toujours impliqués dans toutes les discussions. Cela crée un manque de coordination et une dispersion des efforts. de créer permettra une meilleure coordination des actions, garantira une concertation plus large et aidera à trouver des solutions équilibrées entre la protection des prédateurs et la défense du pastoralisme. Quel est l’avis de la commission

La valorisation de la laine permet aux éleveurs de tirer un revenu complémentaire de la vente des produits de la tonte et de créer une filière de transformation nationale de fertilisants organiques ayant démontré leur pertinence sur le plan agronomique. Outre les débouchés traditionnels comme l’isolation, le matelassage, le paillage agricole et l’habillement, la valorisation sous forme de pellets de laine constitue une méthode vertueuse qui s’inscrit dans une logique d’économie circulaire qu’il est opportun de soutenir et d’accompagner. Les techniques de fabrication de matières fertilisantes issues des produits lainiers sont soumises à la réglementation sanitaire européenne relative aux sous produits animaux (Span) et à la réglementation nationale des supports de culture et de matières fertilisantes. Il semblerait cependant que les États membres n’aient pas tous la même interprétation des exigences techniques définies à l’échelle européenne. Certains pays européens, dont l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, commercialisent en effet des produits interdits à la vente en France. Une fois de plus – et je le déplore –, notre pays a fait le choix

Ensuite, l’article prévoit la possibilité de légiférer par ordonnance pour adapter la nomenclature ICPE et Iota des exploitations en aquaculture. Or les attaques en règle contre la démocratie environnementale et la protection des installations classées

toutes les installations en pisciculture, ce qui est une aberration écologique, une aberration sécuritaire dès lors qu’il s’agit de prévenir le risque d’inondation, une aberration dans la gestion de la ressource en eau, et une aberration pour la préservation même des ressources piscicoles. Nous invitons donc le Sénat à supprimer cet article truffé de régressions environnementales.

Par cet amendement, le Gouvernement propose de supprimer le paragraphe qui vise à exonérer les produits lainiers de l’obligation d’hygiénisation préalable à leur transformation.

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 3 et 4 de l’article 17 qui habilitent le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour adapter le régime concernant, en matière d’aquaculture, les sites classés dans la nomenclature ICPE ou Iota.

Nous proposons de supprimer les alinéas 5 à 9 de l’article 17 visant à exclure les piscicultures de la nomenclature Iota et à leur prévoir un régime d’ICPE dérogatoire au droit commun. Le Gouvernement a engagé des travaux depuis plusieurs mois pour répondre aux besoins des pisciculteurs en matière de simplification de l’encadrement de leur activité, aujourd’hui à cheval sur les deux régimes Iota et ICPE. C’est donc une mesure de simplification majeure qui vous est ici proposée.

Le Gouvernement a engagé un important chantier de simplification en matière d’aquaculture, en particulier pour simplifier les régimes d’activité des

Dans le cadre de ce nouveau régime d’enregistrement, les prescriptions Iota seront instruites au cours de la même demande afin de simplifier grandement la charge de l’exploitant et de lui donner une plus grande visibilité.

un rappel au règlement. Mon rappel au règlement est fondé sur l’article 45 de notre règlement relatif à la recevabilité financière des amendements.

Il a été déclaré irrecevable au motif qu’une extension du droit de préemption est considérée comme une extension des compétences, et donc une charge publique. Cette interprétation me semble erronée, d’autant que les Safer revendront les parcelles acquises à des castanéiculteurs. Le droit de préemption visé par l’amendement déclaré irrecevable se serait substitué au droit de préférence qui prévaut aujourd’hui. En effet, la loi de modernisation de l’agriculture du 27 juillet 2010 a institué un droit de préférence des propriétaires de parcelles contiguës lors de la vente d’une parcelle boisée d’une superficie inférieure à 4 hectares. Or l’application de cette mesure a posé de nombreuses difficultés aux propriétaires vendeurs, aux notaires et aux Safer. Ainsi, un castanéiculteur, propriétaire d’une parcelle contiguë cadastrée en verger, ne peut prétendre au droit de préférence, car sa parcelle est distincte d’un bois, tandis qu’un propriétaire non agriculteur dont la parcelle est cadastrée en bois peut faire valoir son droit de préférence. cet amendement semble donc essentiel pour favoriser l’accès au foncier des castanéiculteurs, en leur ouvrant la possibilité d’acquérir ces parcelles soit directement, soit par le biais du droit de préemption des Safer, sans que s’exerce le droit de préférence. Tout à fait

La délocalisation de l’industrie du textile français et des sites de lavage vers l’Asie, le développement des fibres synthétiques au détriment des fibres naturelles, ainsi que la baisse des prix à l’échelle mondiale ont conduit les éleveurs ovins français à se désintéresser de la laine. Pourtant, celle ci constitue une ressource naturelle pour la confection de textiles, ainsi que pour la construction ou la protection des sols, de sorte qu’elle pourrait être une source de revenu additionnelle pour les éleveurs. La laine est aussi une ressource essentielle à notre souveraineté industrielle. pour réorganiser la collecte et le lavage de la laine, et pour lui assurer des débouchés industriels suffisants, il faut une réflexion globale et des actions de nature diverse. Certes, nous avons constaté que le Gouvernement n’avait pas d’autre stratégie industrielle que la course au moins disant fiscal et social.

en étroite collaboration avec les professionnels de la filière, qui a abouti, le 16 mai dernier, à la restitution des travaux de rédaction d’une feuille de route. La feuille de route existe donc bel et bien et la structuration de la filière est en marche. Je vous propose donc de retirer votre amendement, monsieur le sénateur.

En effet, les étangs piscicoles constituent un atout majeur pour notre souveraineté alimentaire et pour la préservation de nos territoires. Pourtant, cette filière est trop longtemps restée dans l’ombre. La France compte 120 000 étangs et environ 50 000 pisciculteurs pratiquant une pisciculture extensive. Malgré ce potentiel considérable, la production de poissons d’eau douce a chuté de 60 % en dix ans et, comme l’a rappelé M. le rapporteur, 70 % du poisson consommé en France est importé. Cette situation est d’autant plus préoccupante que le développement de l’aquaculture est une priorité européenne et internationale, ce qui a même été souligné par l’ancien haut commissaire au plan, devenu Premier ministre. L’intégration d’une définition juridique des étangs piscicoles était donc une nécessité. Jusqu’à présent ces espaces étaient soumis à une réglementation éclatée, dispersée entre le code civil, le code rural, le code de l’environnement et le code de l’urbanisme. En l’absence de cadre clair et cohérent, les pisciculteurs faisaient face à une insécurité juridique pesante, freinant le développement de leur activité. Grâce à ces articles, nous posons enfin un cadre solide qui permettra de mieux accompagner la filière. Par ailleurs, il est également fondamental de reconnaître les services écosystémiques rendus par les étangs. Ces milieux jouent en effet un rôle clé dans la préservation de la biodiversité, la gestion de l’eau, la captation du carbone et même la réduction de l’empreinte environnementale de notre alimentation. Comme l’ont démontré des travaux scientifiques récents, les étangs fournissent des protéines animales à faibles

le code de l’environnement définit déjà la pisciculture en tant qu’« exploitation ayant pour objet l’élevage de poissons destinés à la consommation, au repeuplement, à l’ornement, à des fins expérimentales ou scientifiques, ainsi qu’à la valorisation touristique

On en vient à se demander si Matignon pilote réellement l’activité du Gouvernement et du soi disant socle commun… Concernant le fond de l’article, nous avons de sérieux doutes sur l’opportunité de confier au département la prérogative de gestion de l’eau. L’échelon intercommunal nous semble le plus approprié, quand ce n’est pas l’échelon communal dans certains cas particuliers de territoires très peu denses.

cet excellent amendement, inspiré de celui de nos collègues députés socialistes. Je rappelle que les Sdage concernent la prévention de la qualité de l’eau, la gestion des ressources en eau, la protection des milieux aquatiques, la prévention des risques et la participation du public. Tous ces éléments sont impératifs, en particulier la participation du public, et le transfert au département ne peut en aucune façon constituer un vecteur d’accaparement de l’eau pour construire des mégabassines, notamment. Quel

vise à insérer la mention de la commune comme acteur principal dans la gestion des compétences eau et assainissement. Il s’agit de répondre à une problématique essentielle faut il confier ces compétences exclusivement aux intercommunalités, ou bien laisser la possibilité aux communes de continuer à les exercer lorsqu’elles le souhaitent et qu’elles en ont les moyens ? Le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale, a insisté sur la nécessité de redonner du pouvoir aux territoires. Cette mesure s’inscrit pleinement dans cette orientation, en garantissant que les communes puissent conserver la gestion directe de ces services essentiels. Le transfert obligatoire aux intercommunalités a suscité de nombreuses résistances parmi les élus locaux, soucieux de préserver une proximité avec les usagers. Il est donc légitime d’adapter la législation en conséquence, en cohérence avec la proposition de loi

qui ne vise que les syndicats mixtes constitués d’un ou plusieurs groupements de collectivités territoriales et départements.

Cet amendement de Mme Loisier vise à concilier la nécessaire préservation des ressources en eau et le maintien d’une agriculture productive dans les aires d’alimentation de captages d’eau potable.

Pour rappel, la directive SUD interdit les traitements aériens, sauf lorsqu’il n’existe pas d’autre solution viable ou lorsque la pulvérisation aérienne présente des avantages manifestes. Or cette technique de traitement, selon les circonstances et productions locales, présente de nombreux avantages : elle réduit la pénibilité ou la dangerosité dans les parcelles escarpées ; elle ouvre à l’exploitation des parcelles non mécanisables vouées à l’enfrichement ; elle parfait la protection de végétaux inatteignables en hauteur par un traitement au sol par atomiseur ; elle facilite la transition vers des produits naturels nécessitant souvent

élargissement des prérogatives de Chambres d’agriculture France, au détriment du ministère de l’agriculture et de l’autonomie des chambres, irait à l’encontre du respect de la démocratie agricole et de l’adaptation territoriale des missions des chambres. C’est d’autant plus vrai

Cette mesure était censée s’appliquer dès 2024. J’ai plusieurs fois rappelé cet engagement, et mon ministère a tenu cette position tout au long de l’examen du budget.

des sols volcaniques ainsi que des besoins réels en azote des cultures locales, et que les techniques d’épandage soient adaptées aux contraintes topographiques et d’accessibilité des parcelles. Rappelons également que la pérennité des filières agricoles de La Réunion est essentielle pour maintenir et renforcer la sécurité alimentaire de l’île. Or cette pérennité implique la prise en compte des spécificités de cette île, qui ne peut être soumise à des normes en tout point identiques à celles qui sont en

jeudi 13 février 2025 : À dix heures trente : Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi portant diverses mesures visant à adapter le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d’agriculture et de la mutualité sociale agricole (texte de